L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Quelle que soit la position que nous ayons pu avoir, les uns et les autres, sur l'organisation de ces jeux, la décision a été prise, et il nous appartient de faire en sorte qu'ils se réalisent dans les meilleures conditions possible. Je crois que l'Assemblée nationale

nous nous sommes aperçus que l'Assemblée nationale tenait beaucoup à une disposition prévue à l'article 17 , selon laquelle un député et un sénateur siégeraient au comité des rémunérations et au comité d'éthique du COJOP, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.

mesdames, messieurs les sénateurs, je reviens de Pyeongchang, où je suis allée soutenir nos athlètes paralympiques. Quelle fierté, quelle émotion de voir Marie Bochet, Arthur Bauchet, Frédéric François, Benjamin Davier

et entraîneurs et tout l'encadrement mêlent leur énergie pour faire rayonner la France. Des années de préparation pour un mois de compétition, mais quelle compétition ! ! Les jeux, ce sont aussi des milliards de téléspectateurs, des millions de spectateurs, des retombées économiques considérables et, plus que tout peut-être, un formidable

tenir les délais ; respecter le budget. Et quand on sait ce qu'il nous faut réaliser, je vous le dis, nous n'aurons pas trop de six ans et demi Ce double objectif a motivé le projet de loi, qui vous a été soumis à la fin de l'année dernière et sur lequel vous êtes amenés à vous prononcer définitivement aujourd'hui. Nous sommes conscients que des dérives ont pu, par le passé, écorner l'image des Jeux. Nous ne voulons pas de cela et nous nous dotons, grâce à ce texte et aux structures mises en place, de tous les garde-fous nécessaires pour respecter nos engagements vis-à-vis du CIO et surtout vis-à-vis des Français. Avec mon collègue Gérald Darmanin, j'ai demandé un rapport d'inspection générale pour vérifier que nous étions sur de bons rails. Certains points d'alerte nous ont été communiqués et, pour une parfaite transparence, je vous précise que nous rendrons public ce rapport au début du mois d'avril. Je saurai prendre les décisions qui s'imposent pour concilier héritage et maîtrise des coûts, après m'être entretenue avec les élus locaux et les acteurs concernés.

Vous avez su, collectivement, enrichir ce texte, tout en préservant ses grands équilibres. Par ailleurs, la commission mixte paritaire a su parvenir à un accord, qui aboutit aujourd'hui à un texte dont nous pouvons être satisfaits. je mesure la frustration qui a pu être la vôtre dans un exercice relativement contraint et dont l'objet était finalement peu sportif. nous avons parlé protection des termes, publicité, urbanisme, sécurité, éthique et transparence, mais pas de sport ! Et parce que je partage cette frustration, je prends un engagement devant vous je prends date pour 2019, afin que nous débattions, ensemble, d'une grande loi « sport et société ». Nous travaillerons de manière concertée et anticipée au développement de la pratique sportive, à la démocratie sportive et à l'éthique du sport.

Enfin, j'en terminerai par un élément d'actualité pour mon ministère : le sport est touché, comme tous les secteurs, par des discriminations et différentes formes de violence. Nous ne fermons pas les yeux et, avant de vous rejoindre, j'ai lancé, ce matin même, une campagne nationale de lutte contre les discriminations, afin de sensibiliser nos compatriotes aux bonnes pratiques et de lutter contre les comportements qui n'ont pas leur place dans le sport et sur notre territoire en général. La parole

le projet de loi portant sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 est le fruit d'une attention collective soutenue et d'un travail constructif, insiste. Je remercie tout particulièrement les rapporteurs de ce projet de loi, notamment Mme Muriel Jourda, ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs qui se sont mobilisés à l'occasion Cet événement sportif revêt tout d'abord un caractère diplomatique, puisqu'il rassemblera 15 000 athlètes, 70 000 bénévoles, 11 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs. À l'heure des replis identitaires, des rassemblements nationaux et des crispations frontalières, la France sera, pendant près d'un mois, la terre d'accueil de 206 comités nationaux olympiques et de presque autant de nationalités différentes. Si l'on estime les retombées économiques de cet événement à un montant de 5 à 10 milliards d'euros pour la région francilienne, la valeur réelle et symbolique de ces jeux en termes d'échanges internationaux et interculturels est quant à elle inestimable. Qui plus est, l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 est l'occasion pour la France de démontrer que les enjeux éthiques, économiques, sociaux et environnementaux, que l'on oppose encore trop souvent, peuvent être conciliés au sein d'un même projet d'envergure internationale. et Territoires a présenté un amendement visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Comité national olympique et sportif français. D'abord retiré à la demande du Gouvernement, l'amendement a été déposé par Marie-Pierre de la Gontrie et finalement adopté lors de la commission mixte paritaire. Je félicite les sénateurs et les députés pour leur persévérance et leur désir d'exemplarité en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous rappelle que moins d'une fonction de direction sur cinq est occupée par une femme dans le monde. Grande cause nationale du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes nécessite de faire preuve de persévérance et d'un certain courage politique. L'aménagement d'infrastructures olympiques est aussi l'occasion de remédier, en partie, à certains déséquilibres territoriaux. À titre d'exemple, la construction d'un centre aquatique en Seine-Saint-Denis, où la moitié des élèves arrive au collège sans savoir nager, donne un sens et une portée sociale aux investissements publics et privés. Je me dois néanmoins de rappeler que les déséquilibres territoriaux s'étendent bien au-delà de la région parisienne. Une question reste en suspens : comment étendre les retombées socio-économiques des jeux Olympiques 2024 à l'ensemble des territoires, y compris aux zones rurales ?

Cette disposition s'inscrit dans une volonté plus large de valoriser les critères de responsabilité sociétale dans les décisions prises par les acteurs publics et privés. Je note qu'un rapport a été remis cette semaine au ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, proposant de changer la définition même de l'entreprise. Enfin, les jeux Olympiques de 2024 seront aussi les premiers jeux paralympiques français. À ce titre, la France devra relever le défi de l'accessibilité des espaces ouverts au public pour les 4 000 athlètes et les milliers de spectateurs concernés. Au-delà de cet événement de quelques semaines, il s'agira bien sûr de trouver des solutions durables d'accessibilité- vous en avez parlé, madame le rapporteur -pour les 12 millions de personnes qui vivent chaque jour, en France, avec un handicap. S'il appartient au Parlement d'offrir un cadre législatif sur mesure pour faciliter l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les attentes de la société en termes de soutenabilité budgétaire, de sécurité et d'exemplarité de la gouvernance sont fortes et légitimes.

Le groupe du RDSE votera d'ailleurs très majoritairement ce texte, qui est nécessaire pour que Paris et la France soient au rendez-vous en 2024. Ce projet de loi ne lève cependant pas toutes les interrogations relatives à la préparation et à l'organisation des Jeux. ces derniers sont nimbés d'une aura presque magique, qui repose sur le sentiment que la ville hôte accueille le monde, le temps de deux quinzaines, olympique et paralympique. Cette mythologie, qui renvoie à l'antique, s'enrichit à chaque olympiade du récit des exploits des athlètes, de Spyrídon Loúis, lointain descendant de Phidippidès, à Martin Fourcade ou Marie Bochet. Je tiens d'ailleurs à féliciter cette dernière, ainsi que les autres athlètes paralympiques, qui écrivent actuellement à Pyeongchang de belles pages de l'histoire du sport français. Cette dimension magique a cependant souvent aveuglé les organisateurs, prêts à tout pour décrocher les jeux, causant des dépassements de budget parfois pharaoniques. Le Gouvernement semble déterminé à se prémunir contre cette dérive, bien aidé, il est vrai, par le fait que la grande majorité des installations est déjà construite. Pour celles qu'il faut encore ériger, le titre II de ce projet de loi vient apporter des assouplissements importants en matière de construction et d'aménagement. L'impératif du respect des délais de livraison justifie des mécanismes dérogatoires au droit commun. Je me réjouis, à cet égard, que la commission mixte paritaire ait maintenu la modification adoptée par le Sénat, visant à encourager les travaux de mise en accessibilité des métros parisien et marseillais. Nous aurons à reparler de ces enjeux dans le futur projet de loi « mobilités Je me réjouis également du maintien, dans la rédaction du Sénat, de l'article 10 relatif à la charte d'insertion et de responsabilité sociale. Je souhaite que la SOLIDEO et l'ensemble des maîtres d'ouvrage intègrent une clause d'insertion sociale et professionnelle dans tous les marchés publics, comme le permet la législation, afin que les grands chantiers olympiques, dont la majorité se situe en Seine-Saint-Denis, puissent bénéficier à ce territoire et à ses habitants. La première partie du projet de loi, qui rassemblait les aménagements législatifs rendus nécessaires par le contrat de ville hôte, a, elle aussi, subi peu de modifications. Telle était la volonté du Gouvernement, même si l'on peut s'interroger sur les conditions qui entourent la conclusion de ces documents fondamentaux et sur certaines clauses exorbitantes. Quelques menues améliorations ont néanmoins été apportées pour encourager la parité au sein du mouvement olympique et sportif français et un compromis a été trouvé en

du groupe du RDSE seront particulièrement attentifs à ce que la représentation nationale soit régulièrement informée de l'état d'avancement des différents chantiers et de l'apparition de nouvelles contraintes. Ils demeureront également vigilants sur le respect des garanties apportées, notamment s'agissant des monuments inscrits ou classés. Le rapport de la Cour des comptes, prévu à l'article 18, et le jaune budgétaire, qui sera annexé aux prochains projets de loi de finances, y contribueront. Et j'ai noté que Mme la ministre a fait part de sa disponibilité pour répondre aux questions des parlementaires. Je regrette néanmoins d'avoir appris, par la voie de fuites opportunes dans la presse, l'existence d'un rapport de plusieurs administrations s'inquiétant de possibles dérapages budgétaires Sa lecture nous aurait sans doute permis de légiférer de manière plus éclairée, alors qu'un montant de 1,5 milliard d'euros d'argent public sera consacré aux jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la ministre, vous accordez également une grande importance à l'impact et à l'héritage de ces jeux. Ils se mesurent à l'aune des retombées économiques à court et moyen terme, mais aussi à celle des transformations apportées à la métropole. Madame la ministre, vous assignez un autre objectif ambitieux à l'horizon 2024, celui d'encourager l'activité physique et sportive de trois millions de personnes. Cet enjeu relève de la santé publique et des politiques d'inclusion. Or, pour atteindre cet objectif, il faudra des infrastructures sportives de qualité sur tout le territoire national et un fort tissu associatif sportif. le développement du sport, le CNDS, nous alerte. En 2018, celui-ci soutiendra moins de projets d'équipement et subventionnera moins d'associations. Et la privatisation annoncée de la Française des jeux, renforce l'inquiétude sur la pérennité de ses ressources. De surcroît, le secteur associatif sportif est particulièrement affecté par la diminution des aides en faveur des contrats aidés. Une autre inquiétude porte sur la diffusion télévisée des jeux Je veux brièvement redire à cette tribune notre attachement à la diffusion « en clair » de la majorité des épreuves. La plupart de nos compatriotes ne verront, en effet, les JO qu'à la télévision. je regrette que l'amendement que nous avions déposé, en première lecture, pour rendre gratuite la retransmission publique d'épreuves par les collectivités et les associations ait subi les foudres de l'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution, selon une interprétation maximaliste. mes chers collègues, je suis convaincue que, pour être belle, la grande fête des Jeux doit irriguer tous nos territoires. Nous avons l'ardente obligation d'inventer un modèle de jeux plus durables, plus sobres, moins mercantiles. Et je ne parle pas du mouvement olympique international, qui aurait aussi besoin d'une vaste réforme. Il faut conclure, ma chère collègue. C'est à cette condition que les jeux Olympiques et Paralympiques seront ceux de toute la France et de tous les Français. C'est à cette condition que ces olympiades seront réussies et exemplaires.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je souhaiterais tout d'abord saluer l'esprit de responsabilité et d'unité qui a animé les parlementaires pour la rédaction du texte final. Cet esprit est à l'image de celui des jeux Olympiques : la coopération et l'union sont la clef de la réussite. Cette réussite, nous l'organisons aussi au travers de ce projet de loi, qui respecte les trois engagements phares

Les articles adoptés en commission mixte paritaire sont le reflet de ces trois volets. Ils sont le fruit de la rédaction aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat et résultent parfois d'un accord entre les députés et sénateurs réunis pour rédiger le texte final. Nous nous en félicitons.

représentation équilibrée entre les femmes et les hommes afin de favoriser la parité au sein du Comité national olympique et sportif. Concernant le texte dans son ensemble, il se divise en quatre titres. Le titre I expose les dispositions relatives aux contrats de ville hôte.

les sites historiques par exemple. Ces mesures transitoires et non définitives, strictement encadrées par le texte, garantissent le respect de nos monuments, tout en permettant la promotion de l'événement et de notre patrimoine à l'occasion de cette manifestation exceptionnelle. Le titre II, relatif à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement, au logement et aux transports, est largement issu de la rédaction adoptée au Sénat. Le travail des parlementaires a ici consisté à simplifier les procédures de mise en accessibilité du métro parisien et marseillais, et ce afin de laisser un « héritage paralympique » en rendant certaines stations accessibles aux personnes en situation de handicap. Là encore, nous ne pouvons que nous féliciter d'une telle mesure, qui, en plus de permettre une organisation adéquate des jeux, engage notre société sur la voie d'un meilleur vivre ensemble. Dans le cadre de cet héritage que doivent laisser les jeux, la commission mixte paritaire s'est aussi accordée sur l'assainissement de la Seine, qui deviendra l'un des bassins olympiques. Les procédures de participation du public à l'aménagement et à la construction des sites olympiques ont aussi été renforcées, ce qui, je l'espère, sera peu à peu généralisé dans nos futurs textes de loi. Suivant l'ordre du texte, j'en arrive au titre III, relatif à la sécurité. L'article 14 du présent titre a fait consensus il autorise la création temporaire, pendant la durée de l'événement, de voies de circulation dédiées aux véhicules de services de secours et de sécurité, ainsi qu'aux personnes accréditées dans le cadre de ces jeux. Cette mesure permettra d'assurer convenablement le bon déroulement des Jeux, mais aussi de désengorger le trafic automobile, sans doute bien chargé en Île-de-France à cette période. Enfin, le titre IV, relatif à l'éthique et à et à l'intégrité, a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, notamment sur les articles 15 et 19. Je salue ici la volonté constructive des parlementaires, qui ont renforcé la lutte contre le dopage en améliorant l'efficacité des sanctions données par l'Agence française de lutte contre le dopage. Concernant la transparence et l'intégrité nécessaires au bon déroulement de ces jeux, l'Agence française anticorruption contrôle désormais non seulement le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi les groupements de collectivités territoriales chargées de recevoir les sportifs et de participer à la construction des sites olympiques. C'est donc un texte cohérent et un symbole de réussite pour le débat parlementaire, capables de participer à l'organisation d'un événement de cette ampleur, qui contribuera au rayonnement national et laissera un héritage bénéfique à nos concitoyens. Il appelle donc un vote unanime de notre part, un vote de cohésion nationale autour d'un projet commun, porteur de sens et de valeurs qui fédèrent notre société.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, aujourd'hui, avec l'adoption de ce projet de loi, nous allons franchir une nouvelle étape indispensable à la réussite du parcours qui nous sépare de la cérémonie d'ouverture du plus grand événement sportif du monde. Nous le faisons avec la conviction que les Jeux de Paris peuvent, si notre pays s'en donne les moyens, devenir non seulement une grande fête mondiale du sport, mais aussi une chance unique pour l'impulsion de pratiques sportives pour tous. Ce second objectif, pour nous central, appellera d'ailleurs d'autres rendez-vous législatifs. Le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui s'en tient pour l'essentiel à la transposition des obligations incombant à la France du fait du contrat signé avec le CIO et le CIP. C'est un passage obligé, une conséquence logique du soutien que nous avons apporté à la candidature. Vous le savez pourtant, nous appelons de nos voeux depuis des années, notamment par la voix de Marie-George Buffet, une réforme internationale des conditions d'attribution des Jeux, notamment pour plus de transparence. Le projet de loi a inclus des dispositions renforcées en matière d'éthique, et nous nous en félicitons. Il a également inclus un article bienvenu encourageant la représentation des femmes dans les instances sportives. Pour notre part, nous serions même favorables à ce que les pays qui interdisent l'accès des femmes à la pratique sportive ne soient plus admis à participer aux jeux. Je souhaite que les Jeux de Paris soient l'occasion d'une belle et grande promotion du sport féminin dans toutes les disciplines. Au-delà de l'adoption de cette première loi, qui ne fait plus débat entre nous, je voudrais une nouvelle fois profiter de l'occasion pour insister sur ce qui nous paraît devoir être mis en chantier rapidement pour un égal accès de toutes et tous, valides et handicapés, à la pratique du sport dans notre pays.

Or les freins à l'accès au sport restent nombreux. Ils sont territoriaux et sociaux, d'abord. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens, souvent jeunes, mais pas seulement, se voient refuser une inscription sportive faute de places, d'encadrement, d'infrastructures suffisantes. À l'école, à l'université, dans l'entreprise, la place et le temps accordés au sport sont indignes d'une grande nation olympique. Nous avons beaucoup de progrès à faire pour résorber les inégalités territoriales en matière d'accès aux équipements, et cela nécessite une ambition nationale.

Ajoutez à cela la partie du matériel non fourni par ces derniers, multipliez par le nombre de personnes pratiquantes dans un foyer et vous arrivez à une charge difficilement supportable pour de nombreuses familles, dans un pays où les salaires et les minima sociaux

budgétaire. Ces freins sont sociétaux, encore, liés à l'éclatement des temps de vie, quand rythmes et horaires de travail conduisent à de nouvelles formes d'isolement social. Comment amener son ou ses enfants ou aller soi-même aux entraînements de fin d'après-midi ou de début de soirée lorsque l'on travaille de plus en plus en horaires décalés, voire le dimanche ? sont culturels, enfin, car les vertus émancipatrices du sport sont refoulées dans notre société, où la marchandisation prend sans cesse le pas sur la fraternité, où la compétition et la performance tendent à l'effacement du au profit la guerre de tous contre tous. D'ailleurs, la question du handisport, qui est très révélatrice de tous ces freins cumulés, devait être une grande cause nationale. Cela nous aiderait à revaloriser la dimension de civilisation du sport pour tous. Si nous croyons réellement à l'ambition d'un véritable héritage sportif des jeux, il faut s'attaquer sans tarder à cette grande ambition, et, je le répète, à la programmation pluriannuelle des moyens nécessaires,

devraient pouvoir bénéficier d'une structure, avec des moyens dédiés. Pour le moment, tel ne semble pas être le cas, et nous le regrettons. Avant de conclure, je formulerai deux remarques encore. L'une concerne les transports. La réalisation pleine et entière du Grand Paris Express est indispensable. Après avoir été tenté par le report du calendrier et des investissements, le Gouvernement a repris des engagements, mais chacun sent bien que la situation reste fragile. Pour tout vous dire, nous ne sommes pas pleinement rassurés et nous restons mobilisés. Si l'on veut que les JO soient une grande fête populaire, ils doivent être un levier pour l'amélioration des conditions de vie et de transport quotidiennes des Franciliens. Je veux redire une nouvelle fois que, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la réalisation de ce grand programme, la réalisation du Charles-de-Gaulle Express, ligne privée inutile et coûteuse, n'avait rien à faire dans ce projet. Plutôt que de séquencer jusqu'en 2030 la livraison des lignes 14 à 18, le Gouvernement a rendu prioritaire ce chantier, et je ne crois pas que cela soit une bonne chose. Ma seconde remarque concerne la question de la diffusion télévisée des JO. des JO. Si l'on veut que l'événement soit une fête populaire, il faut certes permettre une tarification accessible des compétitions- nous apprécions les efforts faits en ce sens -et créer des zones de rencontre, mais il aussi favoriser l'initiative des

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, en 2024, cent ans se seront écoulés depuis que la France a, pour la dernière fois, accueilli les jeux Olympiques. C'est donc avec une certaine émotion et une indéniable fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour voter définitivement le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je tenais de nouveau à saluer le travail accompli par l'ensemble des acteurs du comité de candidature, en particulier son président, Tony Estanguet, ainsi que toutes ses équipes. Les rapporteurs de nos deux assemblées, Muriel Jourda pour le Sénat et Aude Amadou pour l'Assemblée nationale, méritent également d'être félicitées pour la qualité de leurs travaux, au même titre que nos collègues, qui, en commission mixte paritaire, sont parvenus à la conclusion d'un accord, ce dont nous nous réjouissons. Si l'accueil des Jeux de 2024 nous emplit tous de fierté, c'est parce que les jeux Olympiques et Paralympiques sont évidemment bien plus qu'un simple événement sportif international. Ils représentent, dans nos imaginaires collectifs, ce que la compétition sportive a de plus grand et symbolisent un ensemble de valeurs. La responsabilité qui nous incombe était donc lourde, et nous nous devions d'être à la hauteur de cet héritage. À l'aune de ces impératifs, nous avons tenté d'inscrire les Jeux dans un projet à la fois durable et inclusif. Le fait que les collectivités territoriales soient associées à l'élaboration de cette charte est également tout à fait louable, et devrait rassurer les départements. Certains points, toutefois, suscitent toujours autant d'inquiétude. Je pense notamment à certaines réalisations en Seine-Saint-Denis, potentiellement remises en cause par un rapport récent, et, bien évidemment, aux retards du projet Grand Paris Express. L'incertitude la plus totale règne ainsi quant à la desserte de l'aéroport du Bourget par la ligne 17, pourtant stratégique pour les Jeux de 2024. L'hypothèse la plus probable est que les travaux ne seront pas achevés à temps et que la desserte ne sera assurée que par un service de navettes. Cette situation serait tout à fait préjudiciable au bon déroulement de ces jeux et nuirait grandement à l'image de la France en tant que pays hôte. Je ne puis parler des transports sans aborder la ligne 18. Il y a peu, le Premier ministre a annoncé son report en 2030, alors même que cette ligne reliant Orly à Versailles devait permettre de fluidifier le trafic des dizaines de milliers de spectateurs attendus sur les cinq sites olympiques yvelinois. Aussi, permettez-moi de dénoncer ce choix, qui me semble avoir été annoncé quelque peu hâtivement. La France, ce pays, cette vitrine, se doit de rayonner au mieux durant ces journées olympiques. Nous sommes toutefois face à un problème qui se situe en dehors du cadre du présent projet de loi, et qui n'altère en aucun cas la qualité de ce dernier. La question de la participation des territoires est, par ailleurs, loin d'être épuisée, puisque s'ouvrira au printemps le chapitre des bases arrière des jeux. Nos communes pourront alors prendre connaissance des conditions à remplir pour accueillir les équipes sportives et mettre ainsi leurs atouts en valeur. mes chers collègues, pour toutes les raisons précédemment évoquées, le groupe Union Centriste votera en faveur du texte adopté par la commission mixte paritaire, première pierre apportée à l'édifice olympique.

madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà au terme du

le deuxième, plus technique, concerne la modification des procédures d'urbanisme afin de construire dans les temps les infrastructures nécessaires ; enfin, le troisième a a pour objet d'apporter des garanties en matière de déontologie et d'éthique à ces jeux. L'objectif de ce texte est de sécuriser, en amont de 2024, les processus de préparation, afin que cet événement soit une réussite totale sur sur le plan tant de l'organisation que de l'image que nous donnerons de la France au monde entier. Je tiens à saluer la qualité du travail qui a été réalisé en partenariat entre les deux assemblées, sur un sujet qui doit fédérer, au-delà de Paris, l'ensemble des Français.

Enfin, à titre personnel, je suis heureux que l'article 6 du texte adopté par la commission mixte paritaire tienne compte de la modification que j'avais proposée pour mieux valoriser la participation du public. On ne meurt jamais de trop de démocratie Au-delà de cette échéance majeure de 2024, je tiens à rappeler que l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques est un formidable accélérateur des grands projets de la métropole francilienne, projets qui sont aussi d'intérêt national.

donnée aujourd'hui aux visiteurs étrangers arrivant par Roissy et s'aventurant dans les couloirs du RER B. Cette liaison, comme d'ailleurs le Grand Paris Express, figurait dans les atouts mentionnés par la France dans son dossier de candidature aux jeux Olympiques. Et il serait mal venu, admettez-le, que des obstacles, qu'ils soient techniques, juridiques ou financiers, viennent perturber le bon achèvement de cette ligne, qui desservira notamment le village des médias.

la publication du rapport de la Cour des comptes sur les dérapages financiers du projet du Grand Paris Express, puis la gêne du Gouvernement, mis au pied du mur pour tenir ses engagements financiers sur la réalisation dans les délais prévus de ce réseau indispensable pour la survie de la région capitale, ne laissent un dérapage de plus de 13 milliards d'euros, alors même que les travaux sont tout juste entamés, met en doute la capacité de la Société du Grand Paris à tenir ses objectifs, elle qui a été créée justement pour plus d'efficacité. mieux valu confier le projet aux élus franciliens et à Île-de-France Mobilités, c'est-à-dire à l'ex-STIF. Bien sûr, le Premier ministre nous a un peu rassurés en réaffirmant l'engagement de l'État sur la réalisation de ce projet, même si le calendrier a été décalé et l'ordre des priorités bousculé

ligne chère à notre collègue Laure Darcos. Cette ligne ne sera pas réalisée pour les jeux Olympiques, mais elle ne doit pas être sacrifiée. Elle devra impérativement être réalisée en 2027, afin de desservir le plateau de Saclay, futur premier pôle mondial de recherche et d'innovation. Je n'ose pas imaginer les équipes de chercheurs et les investisseurs venus du monde entier sortant à la station RER dénommée Le Guichet- cela ne s'invente pas ! -, pour prendre un bus improbable en direction de Saclay.

au-delà, la pérennisation du dispositif de transports d'une région métropole digne de ce nom. Pour conclure, je tiens à saluer une nouvelle fois la belle unanimité qui a prévalu lors de nos débats, au-delà des clivages politiques. Il est vrai que le sport est, comme toujours, un vecteur fédérateur.

Madame la présidente, madame la ministre, mesdames, messieurs les présidents de commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les discussions relatives au projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ont été riches et constructives. Je tiens à souligner l'oeuvre consensuelle qu'ont pu mener l'Assemblée nationale et le Sénat autour d'un texte d'importance. J'y vois l'illustration des rassemblements possibles des parlementaires, par-delà les affiliations partisanes, autour d'enjeux d'intérêt général. Le texte proposé à l'approbation de notre assemblée respecte l'objet du projet de loi, qui était, d'abord, de transposer au niveau législatif les stipulations du contrat de ville hôte. Le chemin de la réussite matérielle des Jeux de 2024 est ouvert, celui de la réussite éthique également. C'est sur ce sujet que la France innove grandement en mettant en place de nouvelles exigences, qui excèdent les engagements pris devant le CIO. Ce volet démocratique et citoyen prouve très concrètement son utilité. Aux polémiques naissantes touchant au niveau de rémunération des cadres dirigeants du Comité d'organisation, une réponse équilibrée a été apportée.

troisième lieu, la compétence de la Cour des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion des personnes participant à l'organisation des Jeux, ainsi que l'appui de l'Agence française anticorruption, complètent le dispositif d'éthique et de transparence construit autour de ces jeux. Par ailleurs ont été adoptées des dispositions dérogatoires permettant aux et aux partenaires commerciaux de participer au financement. Il me semble que l'équilibre trouvé par le Parlement n'est pas disproportionné entre, d'une part, les besoins financiers visant à couvrir l'organisation et le déroulement de ces jeux et, d'autre part, la protection des sites classés de notre patrimoine national. Ce texte fut aussi l'occasion d'ouvrir des débats que l'inadéquation de ce support législatif ne doit pas masquer. Il en est ainsi de la parité, un sujet essentiel dans le sport, en termes tant de médiatisation que de représentation au sein de ces instances collégiales.

Saluons la simplification des procédures de mise en accessibilité des métros de Paris et de Marseille, qui constitueront des investissements pérennes. De même, grâce à des dispositions impulsées par le Sénat, il sera possible de faire de la Seine un lieu en partage, permettant d'accomplir ce vieux souhait de permettre à nouveau la baignade dans ce fleuve. Il faudra être attentif à l'implantation et au contenu des « camps de base », qui serviront à de nombreux territoires pour profiter de la dynamique enclenchée par les jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L'effet d'entraînement sur l'image du sport devra être mis à profit et articulé de manière effective avec les politiques publiques visant à promouvoir le développement de la pratique sportive. Il s'agit là d'une très belle occasion de soutenir ces politiques de long terme. Les fondations sont là, et je veux souhaiter courage et réussite, pour les travaux à venir, à tous les acteurs de cette magnifique aventure. Les Jeux constitueront un moment majeur pour tous les acteurs politiques, économiques, sportifs, culturels, associatifs et, plus largement, pour l'ensemble des habitants de la région Île-de-France, en raison de la localisation des épreuves et des nouveaux équipements- village olympique, centre de presse, centre nautique -et des infrastructures de transport concernées- bien sûr, je n'oublie pas Marseille pour les épreuves nautiques ! Toutefois, le défi de la mobilisation nationale et territoriale sera à relever, sur la durée. Pour cela, il était déterminant de partir d'un bon pied, et c'est chose faite. L'unanimité du vote sénatorial rejoint l'engouement suscité par le futur événement dans l'opinion publique. Cet engouement est un bien précieux à préserver jusqu'en 2024, afin que les Jeux transcendent le pays d'accueil. Je ne dirai rien sur les soubresauts financiers de dernière minute. Puisque le rapport définitif doit être remis en avril prochain, nous aurons l'occasion d'y revenir. Est aujourd'hui loin dernière nous le funeste 6 juillet 2005, date de la session du CIO qui avait rejeté la candidature de Paris pour 2012. Les conditions permettant de célébrer dignement le centenaire des derniers JO d'été organisés en France- à Paris en 1924 -sont désormais remplies. Ce qui fut perçu ces dernières années comme un passif entre Paris et l'olympisme est aujourd'hui oublié. le chemin fut bien balisé depuis le lancement par Bernard Lapasset, en octobre 2013, d'une étude d'opportunité visant à établir si les conditions d'une candidature de Paris étaient réunies. Tout cela s'est fait grâce à une continuité dans la détermination de l'État, notamment depuis 2013, grâce aux élus locaux concernés, grâce aussi à un parcours plaçant les sportifs sur le devant de la scène et n'hésitant pas à innover. Ainsi, pour la première fois, une organisation non gouvernementale, une ONG- en l'occurrence, de nature environnementale -, est partenaire d'une candidature olympique. En 2024, nous retrouverons, mais démultipliée, l'ambiance de l'Euro 2016. L'impact sur le mouvement sportif- en nombre de pratiquants et conditions de la pratique -, l'accompagnement de la haute performance sportive, l'environnement des clubs, qui font du mouvement sportif le premier mouvement social de France, le mode de vie de nos concitoyens, notamment en termes d'éducation et de santé, les retombées économiques et sociales, y compris en termes d'emplois, l'image et le rayonnement international du pays, la promotion d'une authentique culture du sport dans notre société, l'émotion et la passion en partage seront autant de référents-clés du sens et de l'intérêt de ces jeux. Aussi, paraphrasant le slogan du CNOSF, « le sport, ce n'est pas que du sport », je dirai que « les JO ne sont pas que des JO »

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, j'ai l'honneur d'intervenir en dernier avant le vote définitif du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Comme cela a été rappelé, la commission mixte paritaire est en effet parvenue à la conclusion d'un accord unanime le 20 février dernier, ce dont nous nous félicitons tous. Le présent texte reflète la qualité des débats que nous avons eus au cours des dernières semaines, et le travail de l'ensemble de mes collègues mérite d'être salué. Ce projet de loi, dont les propositions sont principalement techniques, vise à honorer le contrat de ville hôte et constitue, à ce titre, une première étape indispensable. Nous avons cherché, au cours de nos discussions, à créer les conditions les plus favorables au succès des jeux Olympiques et Paralympiques, dans le respect des engagements pris par la France. Cet objectif a, globalement, été atteint, et j'aimerais profiter de mon intervention pour revenir sur certains points. Le premier porte sur la protection accrue des éléments relevant de la propriété olympique et paralympique. Grâce à une étroite collaboration avec le Comité d'organisation, le COJOP, nous sommes en effet parvenus à sécuriser juridiquement ces propriétés olympiques, ce qui devrait rassurer nos partenaires. La France sera indéniablement en mesure de lutter contre les cas de parasitisme et de contrefaçon et, en conséquence, de générer les ressources nécessaires à l'organisation des Jeux, garantissant ainsi la soutenabilité du budget. Je rappelle en effet que l'organisation des Jeux ne pèsera que très peu sur les finances publiques, puisque les ressources des partenariats représentent un tiers du budget prévisionnel. Ce sujet m'amène à l'épineuse question de la publicité. Cette question était sensible et la possibilité d'affichage à proximité des sites et bâtiments classés aura suscité de vives critiques, d'autant plus que les Jeux se dérouleront à proximité, voire à l'intérieur de plusieurs sites protégés. Toutefois, le texte que nous nous apprêtons à voter permettra assurément de concilier ces dérogations publicitaires avec le nécessaire respect de notre patrimoine national. De solides garanties ont été apportées par le COJOP, et les dérogations au code de l'environnement seront, par ailleurs, strictement encadrées. Rappelons aussi que les revenus tirés de l'affichage publicitaire sont absolument nécessaires pour garantir l'équilibre financier des jeux, que nous jugeons tous essentiel. Mes chers collègues, certaines questions relatives à l'organisation des Jeux demeurent néanmoins en suspens. Je pense, premièrement, aux conditions de diffusion des Jeux, évoquées. À ce propos, je regrette qu'il n'ait pas été possible de renforcer dans la loi l'obligation de diffusion en clair pour des raisons de recevabilité financière, ce qui prive les Français de l'accès à de nombreuses épreuves. Aussi, je me dois de plaider la nécessité de trouver un accord entre et les diffuseurs en clair, pour favoriser l'accès des Français à ces

décision importante visant à créer la première étape juridique de la mise en oeuvre des jeux Olympiques. Cette aventure a commencé en 2013, et j'y ai pris toute ma part en tant que ministre des sports. J'ai eu l'occasion, nombreuses reprises, de venir devant la commission concernée de la Haute Assemblée pour présenter ce dossier avec Thierry Braillard. Madame la ministre, la Haute Assemblée vous fait confiance. elle vous demande non seulement de créer les conditions d'un bel écrin- les jeux Olympiques, leur organisation sur le plan juridique, sur le plan matériel et sur le plan des transports -, mais aussi de faire en sorte que cet écrin renferme un beau bijou,

certains orateurs l'ont évoqué, et je salue le travail accompli sur ce dossier par Marie-Pierre de la Gontrie et Jean-Jacques Lozach, qui se sont exprimés -nous souhaitons naturellement que vous obteniez les moyens

Quand on veut un résultat sportif de haute qualité, il faut que la ministre des sports dispose de moyens suffisants ! Je ne sais pas si vous serez encore ministre des sports en 2024. Je vous le souhaite,